Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que le représentant du groupe auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à remercier mon groupe, en particulier son président, François Patriat, d'avoir inscrit ce débat sur la politique familiale à l'ordre du jour et de nous donner ainsi l'occasion de mettre en perspective les différentes réflexions

la mission interministérielle sur la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les allocations familiales, la négociation en cours de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion- la COG -avec la Caisse nationale des allocations familiales et, au niveau européen, la discussion de la proposition de la directive concernant la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Le sujet est donc au coeur de l'actualité sans que, pour autant, le Parlement soit saisi d'un texte. C'est pourquoi le débat d'aujourd'hui est nécessaire pour éclairer la situation actuelle, partager certains constats et identifier des pistes potentielles d'amélioration de notre système. Vous le savez, la politique familiale de notre pays vise aujourd'hui trois objectifs historiques : à sa refondation en 1945, la politique familiale française a eu pour premier objectif le soutien à la natalité par la compensation financière des charges de famille à partir des années soixante-dix, l'accent fut également mis sur le soutien aux familles les plus modestes ; depuis plus de vingt ans, enfin, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle s'est imposée comme un nouvel axe majeur.

les prestations monétaires, les avantages fiscaux et des prestations en nature comme les services publics orientés vers les familles. Le budget que notre pays consacre à la politique familiale est de 59 milliards d'euros

nous faisons davantage que nos voisins Espagnols et Italiens, mais moins que les pays du nord de l'Europe, comme le Danemark. Cette politique familiale forte a porté ses fruits, puisque notre pays connaît, au regard de ses voisins européens, une natalité qui reste soutenue- malgré une baisse depuis 2014 -, une participation élevée des femmes à l'activité économique et une redistribution importante au bénéfice des familles les plus vulnérables. Ce bilan favorable laisse cependant apparaître des marges de progression que je voudrais rapidement évoquer. Tout d'abord, nous devons lutter avec une efficacité accrue contre la pauvreté des familles, notamment monoparentales. Selon l'INSEE, les familles représentaient, en août 2017, 66 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté, à 60 % du niveau de vie médian et s'établit à environ 1 000 euros mensuels. En termes de répartition de la pauvreté selon l'âge, les moins de trente ans représentent 50 % de la population en situation de pauvreté, jeunes ménages compris. S'agissant des seuls enfants, la pauvreté frappe, en France, 19,6 % d'entre eux et 39,3 % de ceux appartenant à des familles monoparentales. Devant ce constat, des mesures pour lutter contre la pauvreté des familles ont été prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 2018 : majoration du montant maximal d'aide auquel les familles monoparentales peuvent prétendre au titre de la garde de leurs enfants par une garde à domicile ou une assistante maternelle, harmonisation des conditions de ressources, des montants de la prestation d'accueil du jeune peut-on s'en tenir là ? La pauvreté des enfants en France reste à un niveau préoccupant, alors que les moyens consacrés à la politique familiale sont considérables. Il faut donc, à mon sens, revoir nos instruments de politique familiale pour les adapter à l'objectif prioritaire de lutte contre la pauvreté des familles. Madame la ministre, la discussion doit s'ouvrir sur l'opportunité de redéployer des dépenses et des avantages fiscaux. Cette question ne se réduit pas, tant s'en faut, à celle de l'universalité

affectent donc près d'un ménage sur deux. Or le maintien ainsi que l'évolution des femmes dans la sphère professionnelle dépendent directement de la capacité de soulager des charges familiales. On observe en effet qu'après l'arrivée du premier enfant, ce sont elles qui, au sein du ménage, passent à temps partiel ou cessent de travailler. Ce bref état des lieux a pour but de nous conduire, madame la ministre, mes chers collègues, à des questionnements variés.

Faut-il envisager l'attribution de l'allocation familiale dès le premier enfant ? Faut-il cibler les jeunes parents, voire attribuer une allocation fixe par enfant ? Comment favoriser l'accès des familles modestes aux modes de garde des jeunes enfants ? Malgré un coût relativement modeste, les modes de garde profitent comparativement peu aux familles dont les revenus sont faibles et dont les difficultés d'insertion les plus fortes. Quelle est la position du Gouvernement français dans la négociation sur la directive européenne, qui vise à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et à encourager un meilleur partage des responsabilités familiales Enfin, au regard des différences qui persistent en la matière entre les départements métropolitains et ceux d'outre-mer, toute prochaine réforme touchant à la politique familiale devra être l'occasion d'un rattrapage pour les outre-mer afin d'aller vers plus d'égalité réelle en termes d'accès aux droits familiaux, en tenant compte des particularités sociales, démographiques et économiques propres à chaque territoire. Tels sont, mes chers collègues, l'état des lieux et les quelques questionnements introductifs au débat de ce jour

Madame la sénatrice, vous avez brossé un tableau très complet de la politique familiale. Nous voyons qu'elle a beaucoup évolué au cours du temps. Elle n'est heureusement pas restée figée, tandis que s'opéraient des changements majeurs dans les conceptions de la famille et dans les réalités que ce terme recouvre. Mais vous avez raison : on peut, on doit aller plus loin. C'est la raison pour laquelle je vous livrerai brièvement ici mes priorités. Je répondrai ensuite aux questions sur des points plus particuliers qui suscitent votre intérêt. votre intérêt. La politique familiale est tout à la fois l'un des piliers majeurs de la sécurité sociale, donc un lieu de démocratie sociale la branche famille, un levier puissant de redistribution au service de la réduction des inégalités de revenus et de conditions d'existence et un vecteur essentiel pour aider toutes les familles à concilier engagement dans la vie professionnelle et vie familiale. Je tiens à l'ensemble de ces objectifs, et il me semble que c'est justement dans leur correcte articulation que se trouve l'originalité de la politique familiale française. Si je suis donc d'accord avec vous, madame la sénatrice, pour dire qu'il faut repenser la politique familiale, je suis également attachée à ses équilibres et je ne prône pas de bouleversement majeur. Plusieurs chantiers mobiliseront en revanche toute mon attention et mes ambitions : le soutien à la parentalité, la promotion de l'intérêt de l'enfant et un meilleur accompagnement des familles au moment des situations de rupture.

Les prestations monétaires, la garde des enfants sont des éléments essentiels, bien sûr, mais il faut aussi des lieux de médiation où échanger sur la fonction parentale, trouver des conseils, exposer ses difficultés sans être jugé. Je ne vous parlerai pas ici de la « maison verte » de Françoise Dolto, mais disons que l'idée est tout simplement de développer ces sortes de lieux qui nous aident à vivre ensemble, parents et enfants, alors que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille Les crèches peuvent et doivent aussi jouer ce rôle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, dans le cadre de la future convention avec la branche famille, de permettre aux personnels des établissements d'accueil du jeune enfant de prendre davantage de temps pour accueillir les parents et échanger avec eux.

Je vais me pencher, avec l'Association des départements de France, sur les missions des services de la PMI et sur les moyens à leur donner pour mieux appuyer concrètement les familles, y compris en allégeant certaines de leurs tâches qui me paraissent aujourd'hui moins utiles. l'intérêt de l'enfant, vous le savez, mon périmètre ministériel comporte la protection de l'enfance en général et l'aide sociale à l'enfance en particulier. Je ne parlerai pas de ce dernier sujet aujourd'hui, mais, sur le premier, il y a sans doute des questions à se poser en ce qui concerne la politique familiale. Celle-ci s'est construite autour d'un objectif louable, qui fait encore aujourd'hui consensus : le soutien à la natalité. Le soutien à la natalité s'intéresse avant tout aux adultes, à leurs contraintes, à leurs soucis, à leurs conditions matérielles d'existence. C'est bien naturel et c'est indispensable, mais l'enfant Bien sûr, en aidant les parents, on aide les enfants, indirectement mais nécessairement ; pour autant, on ne les aide pas « exactement » et pas toujours comme il le faudrait. L'enfant a des besoins propres qu'il faut protéger en tant que tels, auxquels il faut accorder une place. Là encore, je citerai brièvement une référence importante pour moi, Janusz Korczak, que vous connaissez sans doute tous. Il disait qu'il faut se mettre à la hauteur des enfants, c'est-à-dire non pas se baisser, mais s'élever jusqu'à eux, s'étirer, et ce dans un but bien précis : pour ne pas les blesser. Je trouve que ce mot est très juste. Alors je serai attentive à tout ce qui peut blesser les enfants et je chercherai,, à développer ce qui est propre à répondre à leurs besoins fondamentaux : jouer, partir en vacances, apprendre, découvrir. C'est la raison pour laquelle la prochaine convention avec la branche famille et la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté seront fondées sur des axes permettant de porter une attention particulière à ces sujets à travers le soutien à l'apprentissage précoce du langage en crèche et aux activités extrascolaires, extrascolaires, le financement de projets pour les adolescents, par exemple développer une activité de quartier ou soutenir une association par un travail collectif. Ces projets sont parfois minuscules à notre échelle, mais ils ont du sens, parce qu'ils permettent à tous les enfants de s'émanciper, de trouver une place propre, d'agir. Il y a aussi des sujets plus difficiles, notamment celui des violences faites aux enfants, de leur repérage, de leur prévention par tous les acteurs : ceux de la petite enfance, de la santé et de l'éducation nationale. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire en termes de formation, de levée de certains tabous, de travail en réseau pour mieux protéger et éviter le pire. Je recevrai prochainement les conclusions d'un important rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les violences faites aux enfants et j'ai demandé que cette inspection puisse se pencher sur les moyens de développer la prévention en matière de protection de l'enfance. en évoquant la question des ruptures et de leur accompagnement. Vous l'avez dit, madame la sénatrice, notre politique familiale représente des dépenses importantes et remplit correctement ses objectifs. Elle soutient les familles et nous permet un niveau de natalité élevé.

Dans ces moments, la cellule familiale a besoin d'un soutien fort, adapté à ses besoins, rapide. Il faut favoriser la résilience, l'adaptation à ce qui arrive, et aller de l'avant. Il faut des guichets réactifs et souples, un travail en réseau, des aides versées en urgence, des services adaptés. Tout cela, notre système ne le permet pas suffisamment. Ses maux sont bien connus : cloisonnement, démarches inutiles, contrôles superflus. Rien ne les justifie, ni la lutte contre la fraude ni le souci légitime de s'assurer du juste droit. Il s'agit d'un défaut de nos organisations et souvent d'une conception encore assez paternaliste de la solidarité. Je rends ici hommage à la Caisse nationale des allocations familiales pour l'efficacité de ses agents, leur souci de proximité, mais je souhaite que nous allions plus loin l'allégement des démarches,

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la maternité, la parentalité et la prise en charge des personnes en perte d'autonomie représentent les premiers facteurs discriminants dont souffrent les femmes qui sont enfermées dans des emplois à temps partiel et peuvent même être obligées de renoncer à leur travail pour s'occuper de leurs enfants, parfois en situation de handicap, ou d'un proche âgé. En avril 2017, la Commission européenne a proposé d'adopter une nouvelle directive concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Celle-ci, bien inspirée, prévoit une meilleure indemnisation du congé parental et la possibilité de le fractionner, impose un congé paternité de dix jours rémunérés au moins à hauteur de la prestation de maladie, soit le double d'aujourd'hui, et cinq jours de congé rémunéré par an pour s'occuper d'un proche dépendant.

France ! C'est une nouvelle fois l'argument financier qui est avancé par le Président de la République : le grand chantier du quinquennat est sacrifié sur l'autel budgétaire ! Comment s'attaquer véritablement aux inégalités sans une contribution suffisante du budget ? Doit-on comprendre que le Gouvernement se cantonnerait à des mesures cosmétiques pour tendre vers l'égalité des sexes ? Alors que 96 % des congés parentaux sont pris par les mères et seulement 4 % par les pères, nous avons ici une occasion inespérée pour rééquilibrer ce rapport, qui pèse lourdement sur la vie professionnelle et économique des femmes. Madame la ministre, vous savez que l'on touche ici au point nodal de l'inégalité entre les femmes et les hommes de ce pays. L'ensemble des syndicats et des dizaines d'associations vous invitent à franchir le pas et à approuver cette proposition Où est la parité, cette égalité femmes-hommes décrétée grande cause nationale par le Président de la République ? Où placez-vous l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes ? Cette hésitation française est incompréhensible. En 1791, Olympe de Gouges énonçait dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que « la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui proposition de directive, vous pourriez faire honneur à ce principe, en libérant les femmes d'un fardeau héréditaire, et donner un vrai signal politique en faveur de l'égalité réelle. Le Gouvernement va-t-il persister dans son choix de bloquer une réelle avancée sociale, nécessaire aux femmes ? La parole

s'est engagée sur une rémunération de 396 euros par mois pour les personnes qui ne travaillent pas. Nous continuons la négociation avec les différents États membres,

C'est elle qui a soutenu le dynamisme de notre natalité pendant des décennies. C'est elle encore qui a contribué à assurer la pérennité de notre système de retraites. C'est elle enfin qui a accompagné la transformation économique et sociale de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. La baisse constante de la natalité depuis quelques années et la transformation du modèle familial remettent pourtant au coeur du débat public cette question cruciale. Durant le précédent quinquennat, la baisse du quotient familial a été un coup dur porté à un domaine qui doit constituer une priorité ; nous le regrettons.

Madame la ministre, lors de ces débats, vous aviez expliqué que les familles monoparentales allaient bénéficier d'une nouvelle aide à la garde de l'enfant, dite « complément de libre choix du mode de garde », car elles utilisaient moins que les autres familles les crèches collectives, dont les horaires ne sont pas toujours adaptés à leur situation spécifique. Je partage entièrement votre analyse et je pense que ces 138 euros par mois seront une aide effective pour ces familles en difficulté. Mais, au-delà de la question financière, nous savons que décrocher une place en crèche relève bien souvent du parcours du combattant, alors même que les collectivités locales déploient des efforts importants pour développer l'accueil du jeune enfant sur le territoire. Madame la ministre, ne serait-il pas judicieux, dans une démarche de transparence, de mettre en place un barème à points afin d'uniformiser les procédures d'admission et de soutenir plus particulièrement les familles en difficulté ? Nous le savons, accéder aux crèches collectives permet aux parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

sur la proposition de directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des parents et aidants. Depuis plusieurs mois, la France, avec d'autres pays européens, bloque la signature d'un accord sur l'une des dispositions de cette directive : l'harmonisation européenne du congé parental.

La proposition de directive prévoit un alignement de la rémunération du congé parental sur les indemnités maladie, soit 50 % du salaire journalier, ce qui, pour la France, en ferait passer le coût de moins de 400 euros à 950 euros en moyenne. En Allemagne, où l'indemnisation du congé parental est portée à 67 % du salaire net, le taux de recours, pour les pères, est passé de 3 % à 25 % ces dernières années. En Suède aussi, une formule offrant un congé spécifique pour le père et une indemnisation élevée a permis d'augmenter la part des hommes dans le recours au congé parental.

Il s'agit aussi d'une mesure d'harmonisation européenne, harmonisation prônée par le Président de la République. Ce serait la première pierre d'un socle commun de droits sociaux pour l'Europe.

puis dans les Territoires palestiniens, il y a un peu plus d'un an, en janvier 2017, accompagné d'une délégation de sénateurs. J'ai accueilli hier et aujourd'hui la délégation de la Knesset, en présence notamment de notre collègue Philippe Dallier, vice-président du Sénat et président du groupe d'amitié France-Israël, qui, à ce titre, s'est rendu en Israël du 1 au 4 mai avec d'autres membres du groupe d'amitié. Votre venue, monsieur le président de la Knesset, à l'occasion des soixante-dix ans de l'existence de l'État d'Israël, traduit la volonté de renforcer le dialogue entre nos deux institutions, notamment en matière de développement technologique, à deux semaines du lancement de la saison croisée France-Israël. Un colloque a d'ailleurs eu lieu hier matin au Sénat sur le thème : « France-Israël : regards croisés sur l'innovation technologique », », colloque que nous avons ouvert ensemble. Mais votre venue traduit aussi la volonté de renforcer notre dialogue sur un certain nombre de sujets, tels que la culture, l'éducation, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Un accord de coopération interparlementaire- le premier dans l'histoire de nos deux assemblées -a été signé en fin de matinée. L'innovation, l'éducation, les investissements, mais aussi la situation préoccupante au Proche-Orient ont été au coeur de nos échanges. Les événements tragiques intervenus ces derniers jours témoignent en effet d'un regain de tensions lourd de menaces. Toutes les parties doivent faire preuve de retenue et contribuer à la désescalade. Je partage les Je partage les propos tenus par le Président de la République le 15 mai, tout comme ceux qui ont été échangés dans cette assemblée mardi dernier, lors des questions au Gouvernement, sur notre attachement à la solution de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité.

cette quête que l'on ne doit jamais cesser, même dans des temps difficiles et douloureux, lorsque l'on est dans l'obscurité. Au nom du Sénat de la République française, je vous souhaite à nouveau, monsieur le président de la Knesset, ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre délégation,

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, les enfants d'aujourd'hui seront demain les adultes de notre pays : lourde responsabilité pour notre société que celle d'assumer le bien-être d'un petit être en construction psychologique et physique Bien sûr, c'est le rôle essentiel des parents que d'éduquer leurs enfants. Ils n'ont aucune envie d'être dirigés ou contraints en quoi que ce soit dans ce rôle naturel corroboré par l'autorité parentale.

ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ... La vie sociale est devenue compliquée. Les mamans travaillent, les parents ont des difficultés d'organisation de transport, de logement. Ils attendent de l'État

Hélas, beaucoup de couples se séparent et demandent au juge des affaires familiales d'organiser leur désunion, leur séparation et la vie quotidienne des enfants. L'intervention d'une tierce personne est nécessaire pour organiser la garde, alternée ou pas. Si les parents reforment de nouveaux couples, d'autres problèmes peuvent survenir. Madame la ministre, toutes ces évolutions sociales sont très perturbantes quand il s'agit de mener une politique familiale. L'enfant reste-t-il au coeur de toutes les décisions, de ces grands objectifs ?

Les rapports des juges des affaires familiales et des services judiciaires, les médecins scolaires, les centres médico-psychopédagogiques, les services sociaux des départements nous alertent. Le placement, quand l'enfant est en situation de danger avéré au sein de sa famille, peut être envisagé, voire doit être une solution.

Après ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Il a le droit à la tenue d'un entretien professionnel. Nous savons tous ici qu'une longue absence peut être préjudiciable au salarié lors de son retour.

Pour pallier cette inquiétude, après chaque longue absence, un entretien professionnel doit être tenu afin de faciliter la réintégration du salarié et d'éviter son licenciement pour insuffisance professionnelle. En marge de cet entretien, le salarié peut demander une action de formation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail de l'entreprise. Cette demande est aujourd'hui laissée à la libre appréciation du salarié ; cette situation est loin d'être satisfaisante. Ne pensez-vous pas, madame la ministre, que, dans le cadre d'une politique familiale bien pensée, il serait préférable d'aller plus loin, en imaginant par exemple la systématisation d'un temps de reprise en douceur ?

est en baisse pour la troisième année consécutive. Le solde naturel est au plus bas depuis l'après-guerre. Relever ce défi démographique est une nécessité. Les comparaisons internationales soulignent l'existence d'une corrélation importante entre les efforts des États en faveur des familles et le niveau de fécondité.

Pour autant, apporter une réponse plus contemporaine aux difficultés des familles est une nécessité. On pourrait à mon sens envisager deux pistes : le versement des allocations familiales dès le premier enfant,

favoriser les familles les plus pauvres et les familles monoparentales. Nous sommes très attentifs à ce que la branche famille réponde aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui.

et pourtant l'inégalité des chances persiste. La main invisible de l'organisation sociale nourrit les frustrations, les amertumes, que la violence parfois exprime. Elle alimente le caractère héréditaire des classes dominantes et leur entre-soi. Édifiants, les chiffres de fréquentation des crèches, des pratiques culturelles et sportives, des universités et des grandes écoles ! Cela a de terribles conséquences : destins tracés et gâchés, violences, déterminisme social, montée des extrêmes.

aux pratiques culturelles et sportives, des licenciements facilités, dont la perspective fragilise les familles, la remise en cause envisagée de l'accord avec la CNAF sur la scolarisation précoce.

et à surseoir au passage à l'acte, scolarisation à l'âge de deux ans. Bref, il y faut la vision d'une société plus juste et une plus grande détermination. Je rêve que ce débat ne serve pas seulement à cacher les vilains coups de rabot de Bercy, en quête des milliards

Cela exige la création d'un grand service public de la petite enfance. Y êtes-vous prête, madame la ministre ? La parole est à Mme la ministre.

La famille a toujours été, reste et restera la cellule de base de la société. La famille, c'est l'union d'une femme et d'un homme qui ont choisi de vivre ensemble, et c'est ce qui permet la venue au monde d'un ou de plusieurs enfants. C'est la femme qui porte l'enfant, aujourd'hui comme hier et comme demain. C'est ainsi depuis que le monde est monde, et la science, qui permet des avancées dans beaucoup de domaines, ne pourra le changer.

Il serait important que les familles choisissant d'avoir plus d'enfants se voient accorder des indemnités assimilables à un salaire familial, assurant une couverture sociale dans sa globalité

Il appartient aux pouvoirs publics de prendre en compte de l'évolution de la société dans les décisions législatives et réglementaires qui sont prises ; c'est au niveau de la politique familiale qu'il faut agir, et il y a urgence à cela ! La France, comme la plupart des pays occidentaux, connaît un grave problème démographique, lié, dans une large

Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer ce que le Gouvernement propose pour mieux prendre en compte les besoins des familles dans leur fonctionnement au quotidien et créer un contexte favorable à une augmentation de la natalité en France ?

plusieurs observations. Tout d'abord, la complexité de notre système le rend très difficilement compréhensible. Comment expliquer que les enfants de certaines familles ne bénéficient d'aucune aide de l'État, alors que, à titre d'exemple, une famille monoparentale avec quatre enfants perçoit jusqu'à 380 euros par mois et par enfant ? Ensuite, ? Ensuite, les familles françaises sont segmentées en trois groupes : celles qui ont des revenus modestes et perçoivent de nombreuses aides ; celles qui ont des revenus élevés et bénéficient du quotient familial ; enfin, les classes moyennes, qui profitent le moins de ces dispositifs. dispositifs. Conditionner l'octroi de l'aide au fait d'avoir deux enfants et plus est délicat. Premièrement, les conséquences de cette politique sur la natalité ne sont pas facilement mesurables. Deuxièmement, rien ne prouve que les coûts soient croissants en fonction du nombre d'enfants. Troisièmement, il est parfois difficile de définir le rang qu'occupe l'enfant dans des familles recomposées avant le remariage. Madame la ministre, face aux limites

Mesure d'équité, de rationalisation et de simplification, cette AFU se substituerait aux aides familiales existantes, serait versée dès le premier enfant et supprimerait les effets de seuil des prestations familiales. Il me serait agréable, madame la ministre,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, repenser la politique familiale outre-mer est une nécessité. nous connaissons dans nos territoires ultramarins des problématiques statutaires, démographiques, culturelles et sociologiques très différentes, qui nécessitent une politique familiale adaptée à nos particularités.

de plusieurs mois de concertation, de repenser le vivre ensemble en Guadeloupe. Par ce biais, les acteurs de terrain ont pu présenter des idées innovantes et concrètes sur la politique familiale. Ils proposent une nouvelle gouvernance de l'action sociale territoriale, permettant d'ailleurs

devraient, si leurs parents le souhaitent, bénéficier d'un droit de garde. L'idée est donc de mettre en place un dispositif comparable au système du tiers payant, quel que soit le mode de garde retenu par les parents.

dans notre pays et qui faisait, du moins le pensait-on, l'unanimité sur toutes les travées : une politique familiale efficace reposant sur un principe clair, celui de l'universalité de ses allocations. Nous en connaissons les origines, qui remontent au général de Gaulle, en 1945, et la finalité, qui demeure tout à fait actuelle. Quel est le résultat de ce revirement de vos prédécesseurs ? La fécondité moyenne est historiquement en baisse depuis trois ans et vient de passer sous le seuil critique de 1,9 enfant par femme. Pourtant, dans un rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la politique familiale, un député de la majorité préconise d'aller encore plus loin que ce qui a été fait ces cinq dernières années ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre collègue Gilles Lurton, corapporteur Les Républicains, s'en est désolidarisé. madame la ministre, remettre en cause le quotient familial serait une erreur majeure, politique, économique et historique.

Économique, ensuite, à l'heure où notre système de retraite par répartition, qui n'est pas assuré, aux conditions actuelles, pour nos enfants, a toujours besoin de jeunes actifs pour compenser les départs à l'autre bout de la chaîne. Historique, enfin, car plus que supprimer des allocations ou un simple avantage fiscal, ce serait renier une tradition tournée vers l'avenir, qui vise à donner à la France des artisans de sa propre histoire. Madame la ministre, le débat sur la politique familiale ne doit pas se résumer à un prétendu clivage entre conservatisme et progressisme ou entre dogmatisme et réformisme. Ne l'emprisonnons pas dans une fausse lutte des classes, hors d'âge et dépassée, ou dans une politique de compensation court-termiste, mais prenons de la hauteur. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à la plus grande prudence sur ce sujet, au nom des principes de solidarité et de responsabilité qui nous lient vis-à-vis des générations futures. La parole est à

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'évolution démographique à laquelle est confrontée l'Europe tout entière, notamment la France, est sans précédent : baisse des mariages, augmentation des divorces, taux de natalité en berne, taux élevé d'avortements, vieillissement de la population. En France, en 2017, le taux de fécondité s'élève à 1,88 enfant par femme. Nous ne pouvons donc faire l'économie d'une politique nataliste forte et ambitieuse. Pour les familles ayant de jeunes enfants, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle apparaît souvent complexe, notamment pour les femmes, bien sûr. La PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, est un pilier de la politique familiale qui facilite le désir de concilier vie familiale et vie professionnelle. L'allocation contient en effet la prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, enfin le complément de libre choix du mode de garde, qui permet aux parents qui travaillent de financer la garde de leurs enfants. Or votre gouvernement a diminué cette allocation, désormais alignée sur le montant du complément familial. La baisse de la PAJE entraîne une perte totale de 500 millions d'euros pour les familles. Selon l'Union nationale des associations familiales, la PAJE a un rôle certain dans l'augmentation du taux d'emploi des femmes. d'emploi des femmes. Le Président de la République a fait de la défense de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Je vois une contradiction entre cette ambition et la casse de la politique familiale menée par votre gouvernement, dans la continuité d'ailleurs du gouvernement précédent.

de fait majoré de 30 % le complément de mode de garde pour les familles monoparentales, ce qui était un choix stratégique. Nous avons débloqué la prime de naissance qui était gelée dans cette prestation, soit une augmentation de 18,5 euros par mois.

la réplique. Je vous remercie, madame la ministre. La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle doit faire l'objet d'une stratégie globale. Je pense que faire de la politique familiale une variable d'ajustement financier est une erreur.

Elle semble n'être pensée que comme une variable d'ajustement de la politique de redistribution, bien que les deux choses n'aient rigoureusement rien à voir. Surtout, la politique familiale, héritage du Conseil national de la Résistance, se réduit chaque année comme peau de chagrin. Les allocations familiales sont désormais distribuées sous condition de ressources. La majoration de retraite pour les mères de trois enfants et plus a disparu. Il est même question de s'attaquer, cela vient d'être dit, au quotient familial. ne parlerai pas du ministère de la famille, qui, depuis quelques années, joue les Arlésiennes. Le résultat est là, sans appel : le nombre de naissances diminue sans cesse depuis 2015, et l'arrivée à l'Élysée du président Macron n'a pas inversé la tendance, bien au contraire En un mot, la politique familiale, qui fut longtemps une marque distinctive de la France, disparaît rapidement. J'ajoute que, à l'origine, dans les années vingt, après la Grande Guerre, notre politique familiale avait pour objectif d'encourager la natalité en France et la fécondité des Françaises. Aujourd'hui, ce qui reste de la politique familiale est devenu l'une des innombrables pompes aspirantes de l'immigration. Nous le constatons à Mayotte de manière éclatante. Certains ministres et parlementaires de gauche ont déclaré que l'objectif de l'État était d'arracher les enfants à leurs déterminismes familiaux, estimant sans doute que l'État était un meilleur éducateur que les parents. Est-ce pour encourager ce déracinement que vous dites détricoter systématiquement notre politique familiale ? Quoi qu'il en soit, en faisant abstraction des calculs politiciens et des idéologies sectaires, il me semble que, sur l'ensemble des travées de cet hémicycle, nous devrions pouvoir tomber d'accord sur le fait que les parents sont les meilleurs éducateurs pour leurs enfants et que l'État devrait soutenir leurs actions, d'autant que la génération et l'éducation sont les plus beaux investissements que nous puissions faire pour l'avenir du pays. du pays. Il faut conclure ! Madame la ministre, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle direction pour notre politique familiale, afin de mettre l'argent des contribuables français au service de la natalité et de l'éducation des Français, au lieu d'en faire une énième pompe aspirante de l'immigration ou une énième source de financement de l'assistanat ?

Le droit à la retraite issu de ces congés est estimé à 18 milliards d'euros et les dépenses fiscales réalisées le quotient familial sont de l'ordre de 14 milliards d'euros.

je vous remercie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous remercie d'avoir participé à ce débat et à la mise en commun de nos réflexions sur ce sujet primordial et complexe qu'est l'avenir de la politique familiale de notre pays. Ainsi, nous avons pu mettre en lumière de manière élargie à la fois des constats et des visions. De manière pragmatique, il est nécessaire, d'une part, d'évaluer les évolutions des modèles familiaux français et, d'autre part, de considérer les changements de la politique familiale, qui est passée, au fil des décennies, d'une politique purement nataliste à l'accompagnement des ménages sur les thèmes les plus larges : conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, égalité dans la liberté de choix. L'argument nataliste ne doit plus primer. Manque d'études globales, biais temporel entre l'action politique et l'observation éventuelle, effet sur la natalité, il a toujours été difficile d'établir un lien de cause à effet entre les politiques mises en oeuvre et leurs répercussions dans la société. Que la politique familiale ait, jusqu'ici, eu un effet ou non sur la natalité des Français, celle-ci ne suffit apparemment plus à maintenir le seuil de fécondité au-dessus du seuil symbolique et tant recherché de deux enfants par femme. avec près de quatre-vingts ans de recul, la pertinence de l'objectif nataliste de notre politique familiale est à questionner. Les échanges constructifs que nous avons eus nous auront permis de partager un constat large, faisant état de la nécessité de la dimension redistributive de la politique familiale, mais aussi de l'accompagnement des familles au moment des incidents de la vie, du peu d'attractivité du congé de paternité et de la faible reconnaissance des professions dites « familiales ». Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous appuyer sur un modèle familial unique pour construire les politiques familiales de demain. Le nombre croissant des familles recomposées ou monoparentales en est une illustration significative, parmi d'autres. Les familles monoparentales, souvent confrontées à une situation financière précaire, notamment, sont l'une des priorités du Gouvernement. Plus largement, la stratégie de prévention de la pauvreté du Gouvernement a pour ambition de lutter plus efficacement contre la pauvreté des enfants, donc des familles, quelque 20 % des enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Des visions différentes ont également été exposées pendant nos échanges. Elles été exposées pendant nos échanges. Elles alimentent une vue d'ensemble de nos points de vue. La moitié des femmes passe à temps partiel ou bien cesse son activité rémunératrice après l'arrivée du premier enfant au sein du ménage.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

améliore la qualité des produits et stimule l'innovation. Nous savons bien sûr que ce sont des modèles théoriques et que, dans la pratique, les choses ne se passent pas tout à fait comme cela. Au sein d'une économie mondialisée, la concurrence entre les entreprises de différents pays est rendue possible grâce au libre-échange, qui permet de baisser les barrières de l'échange, les obstacles non tarifaires, les normes, par exemple en matière de santé, de sécurité, mais aussi la propriété intellectuelle. Il permet en théorie aux pays de se spécialiser en fonction de leur productivité- c'est ce que l'on appelle l'avantage comparatif -et aux consommateurs d'avoir accès à un large éventail de biens et de services. Le libre-échange a pourtant bien peiné à s'imposer. Après plusieurs siècles de protectionnisme, il a fallu attendre véritablement la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les freins au commerce international soient réduits, à l'exception notable du qui a permis l'unification de l'Allemagne au travers de son unification douanière. La France elle-même a toujours eu un problème avec la mondialisation, considérée souvent comme négative ou dangereuse. Au contraire, les Pays-Bas,

telle que nous la connaissons aujourd'hui a engendré des géants économiques qui opèrent sur les différents marchés du monde. La position dominante de ces multinationales constitue un réel avantage, dont celles-ci abusent d'ailleurs trop souvent afin de restreindre l'accès au marché d'autres concurrents. Le rôle d'une autorité de la concurrence efficace doit être de sanctionner ces pratiques. C'est ce que fait l'autorité de la concurrence française, qui a notamment réussi dans le domaine de l'internet mobile en 2012. la pratique de la commissaire européenne à la concurrence mérite notre considération, puisque celle-ci a prononcé l'une des peines les plus lourdes d'abus de position dominante, avec une amende de 2,4 milliards d'euros infligée à Google il y a à peine un an. Malgré ces avancées, force est de constater que la situation demeure critique. Nous avons encore de grands progrès à réaliser, même si, avec le développement de l'OMC, nous espérions une régulation des flux commerciaux internationaux,

Cette politique peu morale, bien que la morale n'ait pas grand-chose à faire avec ces questions, et ce traitement de faveur s'appuient sur des failles juridiques et posent un double problème : la difficile émergence d'acteurs européens compétitifs et, bien sûr, le manque à gagner pour les États. Nous devons aussi nous pencher sur les subventions étatiques non déclarées. Je pense à la Chine, dont les

long terme. La situation est difficile entre l'Union européenne et ses plus proches partenaires, à savoir les États-Unis et la Chine, dans le domaine de l'accès aux marchés publics.

ouverts. Doit-on considérer que les secteurs d'une économie nationale, y compris ceux qui présentent un intérêt stratégique particulier, doivent être ouverts sans discrimination à la concurrence étrangère ?

en essayant d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires des géants du numérique, qui devrait rapporter entre 3 milliards et 5 milliards d'euros, mais celle-ci est difficile à mettre en oeuvre. Concernant la préservation de nos intérêts stratégiques, l'extension du décret dit « Montebourg » constitue également une avancée positive. Prévue dans le cadre du futur Plan d'action elle obligera les investisseurs étrangers à obtenir une autorisation de Bercy pour investir en France dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, le domaine spatial, le stockage de données, les

Vous l'avez compris, mes chers collègues, beaucoup a été réalisé en peu de temps afin que notre politique de concurrence soit refondée. Le Gouvernement a montré sa volonté de faire évoluer la situation au niveau national et international, mais force est de constater que beaucoup d'obstacles se dressent sur notre route. La question se pose désormais de savoir comment surmonter ceux-ci surmonter ceux-ci pour atteindre notre objectif d'un modèle de concurrence équitable et durable. C'est, je l'espère, ce que nous permettra de clarifier le débat de cet après-midi.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Richard Yung, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour débattre d'un sujet qui est au centre de nos réflexions économiques : la politique de la concurrence, notamment son évolution dans le contexte de la mondialisation de notre économie. La concurrence est une caractéristique intrinsèque de nos économies de marché : sans concurrence, pas de nouveaux entrants, pas de nouveaux produits, pas de mécanisme efficient de formation du prix. Sans concurrence, c'est la logique de la rente qui s'installe. La politique de concurrence ne bénéficie pas seulement au consommateur : quand elle est bien utilisée, elle permet de faire progresser l'économie dans son ensemble, en faisant respecter l'ordre public économique. Comme vous l'avez très bien dit, monsieur le sénateur, ce débat a passionné plusieurs générations d'économistes, et il prend un relief nouveau avec la construction européenne et l'approfondissement du marché intérieur, avec l'irruption de la mondialisation comme fait économique majeur ces dernières décennies et, très récemment, avec certaines décisions d'un grand partenaire commercial de la France. Permettez-moi de commencer par cette actualité récente. Le 8 mars dernier, le président Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane additionnels sur les importations américaines d'acier et d'aluminium pour des motifs de protection de la sécurité nationale. L'effet de ces mesures va essentiellement se faire sentir sur les alliés des États-Unis, qui sont les principaux fournisseurs de ce pays dans ces deux secteurs : l'Union européenne, mais aussi le Brésil, le Canada, l'Argentine, le Mexique ou la Corée. L'Union européenne a instantanément fait valoir une position ferme, par la voix de la Commission, avec le plein soutien de la France et, unanimement, de tous les États membres. Certes, nous savons que des surcapacités existent dans ces secteurs, mais nous n'en sommes pas l'origine. En outre, l'Europe est un allié des États-Unis et non une menace pour leur sécurité. En tout état de cause, des mesures unilatérales prises par un État en contradiction avec les règles de l'OMC ne sont pas une solution à un problème d'ordre structurel. L'administration Trump a accepté une exemption temporaire de plusieurs États, dont l'Union européenne, qui a été renouvelée le 30 avril, jusqu'au 1 juin prochain. l'Union européenne reste ferme et demande aux États-Unis une exemption permanente et inconditionnelle des mesures sur l'acier et l'aluminium, car nous refuserons, bien sûr, toute négociation commerciale sous la menace. Parallèlement, nous nous sommes mis en capacité de répondre, conformément au droit de l'OMC, aux mesures qui seraient éventuellement mises en oeuvre par les États-Unis, à la fois par la saisine de l'organe de règlement des différends à l'OMC, la mise en place de mesures de sauvegarde pour protéger l'industrie européenne de l'acier de l'acier et des mesures de compensation sur des produits américains ciblés. Enfin, et c'est très important, nous restons ouverts à un dialogue avec les États-Unis sur le futur de l'OMC et sur un renforcement des règles de concurrence mondiale, en particulier sur le contrôle des subventions industrielles. Voilà une illustration concrète, qui continue de fortement mobiliser le Gouvernement, des enjeux mondiaux de la concurrence dans le commerce international. Plus généralement, la France considère que les règles du commerce mondial, telles qu'elles résultent des accords fondateurs de l'OMC datant de 1994, ne répondent que partiellement à la situation d'aujourd'hui. Le fait que certains membres de l'OMC continuent de développer des politiques industrielles reposant sur des systèmes de subventions massives et d'avantages considérables donnés à leurs entreprises nationales constitue bien sûr l'un des principaux défis posés à la compétitivité de nos entreprises et de nos économies. Nos entreprises ne luttent pas toujours à armes égales. Il est donc nécessaire de lutter collectivement contre les surcapacités et de discipliner bien davantage, au niveau multilatéral, les pratiques de subventions massives développées et amplifiées ces dernières années années par certains États. Les surcapacités concernent potentiellement de très nombreux secteurs, y compris des secteurs de haute technologie industrielle, comme les batteries automobiles. Le cadre multilatéral est alors indispensable. Le renforcement des disciplines multilatérales dans le cadre de l'OMC est un enjeu prioritaire sur lequel l'Union européenne, les États-Unis, mais également les puissances émergentes et les pays en développement doivent travailler ensemble. Par ailleurs, la construction d'une « Europe qui protège », voulue par la France, appelle des instruments européens robustes en matière commerciale, car l'Union européenne doit non seulement contribuer au renforcement des règles multilatérales, mais également renforcer ses propres instruments dédiés à la protection de ses intérêts légitimes, dans le strict respect des règles de l'OMC. Or nous avançons : l'Union européenne vient d'adopter une réforme de ses instruments de défense commerciale, dont les deux principaux piliers sont en train d'entrer en vigueur. La nouvelle méthode antidumping de l'Union nous permettra de maintenir des instruments de protection justes et proportionnés, mais parfaitement efficaces pour contrer les pratiques commerciales déloyales. De plus, l'Union s'apprête à publier une réforme de « modernisation des instruments de défense commerciale », qui permettra de renforcer l'arsenal de défense européen. Ce dernier sera rendu plus efficace, plus réactif et plus transparent. D'autres projets méritent d'être signalés pour rétablir des conditions de concurrence équilibrées le règlement sur l'examen des investissements étrangers en Europe, le règlement relatif à la mise en place d'un instrument de réciprocité dans les marchés publics et l'instauration d'un « procureur » commercial européen. notre politique de la concurrence ne doit pas seulement se contenter de s'adapter à la mondialisation. Elle doit aussi répondre aux nouveaux défis que représentent les acteurs du numérique. Vous avez mentionné, monsieur Yung, le cas emblématique des GAFA. Ces nouveaux acteurs, tout en ayant pu stimuler la concurrence et répondre aux attentes des consommateurs, requièrent de nouvelles approches. Nous avons appelé de nos voeux une initiative européenne pour tenir compte de cette économie des plateformes. D'une part, le marché unique numérique reste, à ce stade, dominé par des acteurs extraeuropéens, ce qui implique que l'Europe doit résolument adopter une stratégie offensive afin de permettre l'émergence d'acteurs européens leaders. D'autre part, sur certains marchés de plateformes, l'existence de dysfonctionnements majeurs fortement préjudiciables à l'efficacité des marchés concernés a été mise à jour. Dans ce contexte, il importe d'appréhender au mieux les relations contractuelles entre acteurs économiques du numérique, notamment pour protéger les PME face aux incontournables mastodontes du marché. Notre droit français des pratiques restrictives de concurrence est en pointe pour appréhender certaines pratiques des acteurs du numérique, à l'instar de celles de la grande distribution. Sur ce fondement ont été condamnées les sociétés Booking et Expedia, pour des pratiques déloyales à l'encontre des hôteliers français. Nous avons assigné, avec Bruno Le Maire, Amazon, Google et Apple pour pratiques commerciales déloyales liées au fonctionnement des places de marché ou aux magasins d'applications. Nous plaidons pour que l'Union européenne se dote, elle aussi, d'un cadre juridique adapté. Il faut saluer l'initiative de la Commission européenne de proposer un règlement européen qui mettrait en place un encadrement renforcé des plateformes numériques en Europe. Par ailleurs, vous le savez, la France porte avec beaucoup d'énergie le débat sur la fiscalité, qui est bien évidemment un enjeu majeur de régulation de l'activité des GAFA. Les géants du numérique paient peu ou pas d'impôts dans la plupart des États où ils déploient leur activité et réalisent des bénéfices. Cette situation pose un problème d'équité et mine le fonctionnement du marché intérieur. À cet égard, la proposition de la Commission de taxe sur les services du numérique a permis d'engager la discussion très concrètement avec nos partenaires européens.

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé. Dans le

chers collègues, depuis que l'Europe est l'Europe, la politique de concurrence est inscrite dans son ADN économique. Le traité de Rome, à l'origine de la Communauté économique européenne, prévoyait déjà, en 1957, que la politique de concurrence est une prérogative communautaire. C'est ainsi que, depuis plus d'un demi-siècle, les autorités européennes travaillent à offrir aux citoyens européens la meilleure gamme de produits au meilleur prix, à l'appui d'un environnement concurrentiel pour les entreprises. Le secteur de l'économie numérique ne peut échapper à cette mise en concurrence. Aujourd'hui, en raison des effets de réseaux, quelques grands opérateurs dominent le marché européen : les GAFA- Google, Apple, Facebook, Amazon -et les NATU- Netflix, Airbnb, Tesla et Uber -sont installés sur le marché et freinent l'entrée des PME et des TPE. De nombreuses professions traditionnelles craignent en effet que leur entrée sur le marché du numérique et leur transformation digitale ne les fassent disparaître à très court terme du marché. Les pouvoirs publics ne sont pas pour autant démunis face à cette situation. En 2015, quatre économistes du Conseil d'analyse économique publiaient une note intitulée, faisant état de plusieurs propositions pour ouvrir le secteur de l'économie numérique à la concurrence. Évolution des réglementations en vigueur, soutien aux expérimentations pratiques, ouverture J'ai conscience que vous avez

Comme je le disais, le numérique ne doit pas faire exception ; il doit y régner de bonnes pratiques de concurrence. Nous ne devons pas laisser prospérer des situations anormales d'abus de position dominante ou de rentes de situation, préjudiciables aux nouveaux entrants, à l'innovation et,, à notre économie. Au niveau national, j'ai évoqué l'action du Gouvernement, en particulier les condamnations des sociétés Booking et Expedia, ainsi que les procédures lancées contre Amazon, Google et Apple pour des pratiques commerciales jugées déloyales. Au niveau européen, de récentes décisions ont également confirmé la mobilisation de la Commission européenne, notamment celles contre Google ou contre Apple. Pour autant, nous devons continuer à renforcer notre arsenal juridique, et cela passe d'abord par le rétablissement d'une juste concurrence fiscale. C'est tout l'objet des orientations que nous poussons au niveau européen, avec Bruno Le Maire, pour une juste fiscalisation des GAFA. Il existe une initiative de la Commission européenne, que le Gouvernement soutient très fortement, vue de proposer un règlement européen en faveur d'un encadrement renforcé des plateformes numériques en Europe. La France a été précurseur en la matière, notamment avec la loi pour une République numérique. Il convient de porter ces avancées au niveau européen, pour rééquilibrer les rapports de force entre les plateformes, parfois monopolistiques, et les fournisseurs de ces dernières. Enfin, nous devons poursuivre la réflexion sur les critères autres que le chiffre d'affaires pour l'examen des concentrations, afin de capter certaines transactions dans le domaine du numérique, du type du rachat de WhatsApp par Facebook. Certains États membres, comme l'Allemagne ou l'Autriche, ont déjà fait évoluer leur réglementation en la matière, et nous avons nous-mêmes des réflexions en cours à ce

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pas une semaine ne passe sans que la politique de concurrence dans l'économie mondiale soit sous le feu de l'actualité, en ce sens qu'elle est souvent utilisée comme un outil pour déployer des politiques publiques ou subordonnée à des décisions géostratégiques. Par ailleurs, la définition de la politique de concurrence varie d'un État à l'autre, voire d'un continent à l'autre, et affecte les entreprises publiques et privées, ce qui rend l'approche tout particulièrement délicate et a nécessairement des conséquences sur les stratégies d'implantations industrielles et commerciales. L'équilibre à trouver entre, d'une part, la lutte contre le protectionnisme parfois clairement affiché de certains États, l'entente ou la concurrence déloyale, que vous avez vous-même évoquée, madame la secrétaire d'État, et, d'autre part, l'intérêt des consommateurs et la liberté d'entreprendre est un exercice complexe, qui, certes, ne peut déboucher que sur des résultats imparfaits. À ce jour, quelques bassins géographiques au sein d'organisations régionales connaissent de longue date ces situations ou prennent des initiatives louables pour concilier ces impératifs avec des règles particulièrement transparentes. Je pense bien entendu, en premier lieu, à l'Union européenne, qui a fait de la politique de la concurrence un pilier de sa construction. Il ne faut pas cependant que cet effort éthique de la France et des pays de l'Union européenne cède à une forme de naïveté, qui ne ferait que pénaliser nos économies et empêcher la constitution de champions européens, dont l'émergence est particulièrement souhaitable dans le cadre d'une concurrence mondialisée. Ma question portera sur la manière d'aborder, sur le plan éthique et sur le plan opérationnel, de graves atteintes au droit légitime des entreprises de librement commercer face à des décisions de boycott décrétées de façon unilatérale par certains pays. Je pense en particulier à des pays dits « amis », comme les États-Unis, qui veulent empêcher toute entreprise d'entretenir des relations d'affaires avec l'Iran, et ce au mépris de l'ensemble des règles internationales, puisque leurs décisions politiques et économiques ont un caractère totalement unilatéral. Quelle réponse apporter à cette difficulté majeure, qui, en dehors de son caractère néfaste sur le plan géopolitique et en termes de sécurité, est la manifestation d'une attitude impérialiste et constitue une entrave insupportable à la liberté du commerce et des échanges ? La parole est à Mme la secrétaire

L'Europe doit affirmer sa souveraineté économique. Pour cela, nous allons travailler sur trois pistes. Premièrement, il convient de renforcer les outils existants pour empêcher l'application de lois extraterritoriales extraterritoriales et protéger nos entreprises. S'il existe un règlement européen de blocage, publié en 1996, celui-ci n'est pas parfait et doit donc être révisé, renforcé, afin d'inclure les dispositions sur l'Iran. il importe de créer les moyens de notre autonomie financière, car le financement de nos entreprises et de leurs investissements dans cette zone est le nerf de la guerre. Nous devons donc mettre en place des instruments de financement européens quand les canaux traditionnels ne peuvent plus être utilisés. Troisièmement, et enfin, il nous faut nous donner les moyens de parler d'égal à égal avec les États-Unis, en particulier avec l'OFAC américain, le bureau qui fait partie du Trésor, met en oeuvre les sanctions et poursuit les entreprises. Nous réfléchissons à la création d'un OFAC européen. En un mot, nous devons nous donner les moyens, en Europe, de façon autonome, de pouvoir continuer à commercer avec les pays et dans des conditions que nous estimons légitimes. La parole

Bizet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la politique de concurrence est une dimension historique fondamentale de la construction européenne depuis les années Seule une concurrence libre et non faussée permet au marché unique de fonctionner efficacement et de produire pleinement ses effets, qu'il s'agisse de la dynamisation des entreprises, de l'accroissement de la compétitivité ou de la baisse des prix pour les consommateurs. Or nous sommes aujourd'hui confrontés à plusieurs défis : tout d'abord, l'accélération des évolutions de l'environnement économique international ; ensuite, l'émergence de nouveaux acteurs, dont les pratiques sont parfois discutables au regard des principes de concurrence ; enfin, le développement des échanges matériels et immatériels. Autant d'éléments qui doivent conduire l'Union européenne à adapter sans plus tarder sa politique de concurrence. l'exemple de son approche en matière de contrôle des concentrations d'entreprises. Vous le savez, trop souvent, nos entreprises sont empêchées de se rapprocher de partenaires européens dans des secteurs-clés. Elles sont condamnées à rechercher des alliances extraeuropéennes. C'est la condition pour atteindre une taille critique qui leur permette d'affronter la concurrence internationale. L'Europe perd ainsi le contrôle des technologies qu'elle a elle-même créées. Elle devient dépendante des centres de décision étrangers ; sa souveraineté économique est fragilisée. Voilà tout simplement mise en cause une approche datée, restrictive, d'une politique de la concurrence, qui doit changer d'échelle de référence. La commission des affaires européennes du Sénat le répète depuis longtemps, cessons d'être naïfs, cessons de mettre en oeuvre une vision inadaptée du marché pertinent. Cette approche erronée empêche l'émergence de champions européens capables d'affronter la compétition internationale. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire comment le Gouvernement entend faire évoluer les approches européennes en la matière, dans un domaine qui relève de la compétence exclusive de l'Union ? Au-delà, quelles sont les perspectives de rééquilibrage de la concurrence au niveau international, alors que des États interviennent directement au soutien de leurs entreprises nationales, tant en matière d'investissements directs étrangers qu'en matière d'offres de service ? Et je ne ferai que mentionner la dimension anticoncurrentielle de l'application extraterritoriale des lois américaines ; ce sujet mériterait un débat à lui tout seul. Très bien

Le Gouvernement a montré d'ailleurs qu'il était prêt à l'action, à l'occasion d'opérations récentes de rapprochement. C'est un sujet que nous continuerons à porter dans le cadre de la promotion d'une politique européenne industrielle.

les instruments de défense en matière de politique commerciale sont renforcés et rendus plus efficaces, plus réactifs et plus transparents. Nous continuerons à soutenir des mesures allant dans le sens d'un renforcement des instruments de défense commerciale, notamment en poussant à l'adoption du règlement règlement sur les investissements étrangers au niveau de l'Union européenne, à l'adoption d'un règlement relatif à la mise en place de la réciprocité dans les marchés publics et à l'instauration du procureur commercial européen. Au niveau national, notre arsenal en matière de contrôle des investissements étrangers va également être renforcé dans le cadre de la future loi PACTE, comme l'a annoncé le Premier ministre : davantage de secteurs seront soumis à la procédure de contrôle, et les sanctions prononcées seront plus crédibles et efficaces. La parole

nous parlons de « concurrence libre et non faussée », objectif inscrit dans le préambule du traité fondant la Communauté économique européenne. On ne peut nier, plus de soixante ans après, les retombées positives de cette vision économique. Pour autant, il existe des territoires français, européens, restés à l'écart, qui, eux aussi, rêvent de prospérité et attendent leurs « trente glorieuses ». Les territoires ultramarins, puisqu'il s'agit d'eux, restent coincés dans une dépendance économique quasi exclusive avec la France ou l'Union européenne, à l'écart de leur environnement régional. En effet, si l'accord de Cotonou, adopté en 2000 entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique- les pays ACP -, donne à ces pays un large accès préférentiel au marché de l'Union européenne, 92 % de leurs produits y entrent en franchise de droits de douane, cet accord est asymétrique, sans réciprocité. Conséquence : les entreprises ultramarines se retrouvent concurrencées par des produits issus des pays ACP bénéficiant des mêmes conditions d'accès au marché européen, souvent subventionnés par l'Europe, fabriqués selon des normes sociales et environnementales beaucoup moins contraignantes, sans pour autant voir en contrepartie s'ouvrir à elles de nouveaux marchés. Nous sommes donc arrivés à un paradoxe, dans lequel l'Europe, partant d'une volonté louable de faire de l'aide au développement fondée sur le commerce et la libération des échanges, a organisé une concurrence déloyale et complètement faussée au détriment de nos outre-mer. Personnellement, j'ai vu s'effondrer la riziculture en Guyane, soumise à la réglementation européenne et française, quand, dans le même temps, à quelques kilomètres de là, elle se développait au Suriname. Aujourd'hui, vous trouvez du riz du Suriname dans tous les supermarchés européens, alors que le riz de Guyane a disparu. Madame la secrétaire d'État, l'accord de Cotonou arrive à son terme en février 2020 et les négociations entre l'UE et les pays ACP doivent commencer, au plus tard, en août de cette année. Pouvez-vous nous assurer que, cette fois, les régions ultrapériphériques ne seront pas les laissés-pour-compte de ces négociations ?

de l'accord de Cotonou, qui structure la relation entre l'Union européenne et les pays ACP et qui prendra fin en 2020. Ce mandat porte sur la négociation, par la Commission, du futur accord de dialogue politique avec les pays ACP. Dans le cadre des discussions sur ce mandat, la France se montre attentive au traitement des régions Caraïbes et Pacifique, au sein desquelles la présence de pays et territoires d'outre-mer et de régions ultrapériphériques constitue une opportunité pour l'UE de consolider une approche régionale du développement. Les autorités françaises ont proposé que les territoires ultramarins et les régions ultrapériphériques soient associés à la mise en oeuvre de l'accord et que des modalités spécifiques soient prévues pour le développement de projets de coopération conjoints

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie le groupe La République En Marche d'avoir proposé l'organisation de ce débat. Il est en effet intéressant de nous interroger sur notre politique de concurrence, qui mérite peut-être mieux que des mesures de fiscal, telles que la suppression envisagée de l'. du paradigme concurrentiel mis en avant par le Gouvernement, je souhaiterais évoquer un autre paradigme qui devrait recueillir toute votre attention : je veux bien sûr parler d'environnement, madame la secrétaire d'État. C'est un domaine souvent évoqué par le Président de la République dans ses discours, mais dont on peine à voir les réalisations concrètes. Les récentes interrogations du ministre de la transition écologique et solidaire sur la feuille de route écologique du Gouvernement démontrent que le « nouveau monde » ne sera pas si vert, si ce n'est de façade. Par exemple, les accords internationaux de libre-échange risquent d'entraîner une harmonisation par le bas des normes environnementales. Où en est-on, madame la secrétaire d'État, du projet de « veto climatique », qui permettrait d'empêcher des intérêts privés supranationaux de contourner la loi en matière d'obligations environnementales ? les tribunaux d'arbitrage, chargés de régler les différends entre États et investisseurs, peuvent être un instrument dévastateur pour nos législations. Regardons la réalité en face. Ce veto, très attendu par la société civile, garantirait la primauté de l'accord de Paris sur le climat sur d'autres accords internationaux, tels que le CETA et, demain, le Mercosur. Où en sont les négociations européennes sur ce veto climatique, que Nicolas Hulot défendait à l'automne dernier ? Dans le climat de guerre économique actuel, François Mitterrand, de « guerre sans mort, mais de guerre à mort », quelles sont les options choisies par le Gouvernement pour faire du développement soutenable ou durable

environnementaux que nous nous fixons. C'est bien un débat qui a émergé au moment de la signature de l'accord CETA et qui a amené le Gouvernement à prendre des positions très en pointe s'agissant des objectifs, sur le fait fait que les valeurs environnementales et les objectifs environnementaux de l'Union européenne doivent être pleinement reflétés dans sa politique commerciale et dans les futurs accords qui seront négociés Sur ce sujet, je puis vous assurer que nous travaillons avec la Commission européenne et que nous poussons cette idée, largement reconnue.

l'État, sous l'impulsion européenne, a laissé notamment libre cours au social. Ainsi, dans les entreprises industrielles, de nombreuses restructurations ont eu lieu ; la valeur du travail a été niée, au profit de la rémunération de l'actionnariat privé. Les délocalisations et les licenciements boursiers se sont multipliés, alors que l'État devrait les interdire. Il nous paraît essentiel de renoncer au dogme, aujourd'hui infondé, de la concurrence libre et non faussée. La concurrence n'est pas la seule loi naturelle du marché. La réglementation et la régulation lui sont tout aussi nécessaires. En effet, les échanges marchands ont gagné une telle ampleur qu'ils ne répondent plus aux besoins humains et ne favorisent que des gains financiers déconnectés de l'économie réelle. C'est pourquoi il est impératif de respecter et de revaloriser nos services publics, voire de réaffirmer la notion de service public à la française, comme le droit de l'Union européenne nous y autorise. Cela implique de protéger les infrastructures essentielles, de reconnaître que certains biens et secteurs- énergie, transport, santé, éducation, la liste n'est pas exhaustive -sont non pas des marchandises, mais des biens communs de l'humanité. Or la Commission européenne a négocié un nombre important d'accords de libre-échange avec des partenaires extérieurs. Loin de mettre en avant des clauses de réciprocité sociale et environnementale, ces accords tendent à niveler par le bas nos standards nationaux et européens. Dès lors, une question se pose ces différents accords servent-ils pleinement les intérêts des citoyens et des entreprises ? D'un point de vue juridique, une politique de concurrence doit s'appuyer sur un réseau de contrôle efficace sur tout le territoire, sur un renforcement des moyens et des compétences de la répression des fraudes. Il doit aussi renforcer le droit de la concurrence dans son volet répression. le mouvement de dépénalisation du droit des affaires et du droit de la concurrence fragilise le rôle de l'État, gardien de l'ordre public économique. Une politique de concurrence doit savoir protéger les entreprises,

Le Président de la République a d'ailleurs insisté sur la nécessité de ne pas faire preuve de naïveté en matière de concurrence. Cette approche, qui vise à garantir la coexistence entre les mécanismes de marché et les activités économiques d'intérêt général, est une constante historique de notre action européenne. La France a toujours promu ce modèle, qui préserve les services publics, et elle a plutôt réussi, le droit européen de la concurrence s'étant largement inspiré du droit français.

et routières, l'ARAFER, pour réguler le marché du transport par autocar, avec comme souci de préserver la qualité et la continuité du service public. S'agissant du rôle de l'État comme régulateur et garant

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les accords commerciaux entre l'Union européenne et un certain nombre de pays- Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil -posent le -posent le problème de l'harmonisation et de la cohérence des normes et principes sociaux, sanitaires et environnementaux auxquels les produits agricoles sont soumis. soumis. Des contraintes importantes sont aussi une garantie de qualité des produits agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, l'agriculture française ne peut lutter face à la concurrence internationale, voire européenne, qui applique des normes sanitaires et environnementales très éloignées de notre réglementation. Les produits agricoles correspondant à l'exigence des consommateurs sont des produits

votre réponse, madame la ministre,

Par ailleurs, les ouvertures des marchés extérieurs obtenues en retour doivent être substantielles, afin de garantir l'équilibre des accords.

Enfin, les normes et les standards européens, notamment en matière de protection des indications géographiques, doivent être promus. Ces négociations commerciales doivent nous permettre d'exporter notre modèle, nos niveaux d'exigence et nos indications géographiques, afin que ceux-ci soient aussi mieux protégés à l'extérieur. En effet, les avantages et les gains potentiels des négociations commerciales pour nos filières agricoles sont substantiels, en ouvrant de nouveaux marchés pour nos exportateurs. Prenons l'exemple de la viande bovine : nous avons des intérêts défensifs à l'égard de certains partenaires, et non des moindres, et non des moindres, mais aussi des intérêts offensifs vis-à-vis d'autres partenaires tout aussi importants. Les négociations menées par l'Union européenne dans le cadre d'accords de libre-échange ou les négociations bilatérales sanitaires menées par le gouvernement français devraient ainsi permettre, dans les années qui viennent, l'ouverture de marchés asiatiques comme la Corée du Sud Sud ou la Chine, avec la levée effective de l'embargo ESB annoncé par les autorités chinoises lors de la visite en Chine du Président de la République. Je pourrais aussi citer des exemples de marchés ouverts sur le fromage.

que le souci de l'empreinte carbone et de la lutte contre le changement climatique soit partagé par un maximum de pays.

La politique de concurrence au niveau mondial nous amène à nous interroger sur les questions de concentrations d'entreprise et sur les régulations internationales qui peuvent intervenir. Les phénomènes de concentration sont récurrents et touchent quasiment tous les secteurs de l'économie. Pour leurs promoteurs, ils sont favorables, non seulement aux entreprises, avec des capacités nouvelles de levées de fonds et des effets de mutualisation, mais aussi aux consommateurs, par une diminution des prix. Ces concentrations conduisent toutefois à des situations de monopole, et les craintes s'amplifient actuellement dans un certain nombre de domaines. Je pense notamment aux entreprises du numérique et de l'internet, qui détiennent énormément de données personnelles. Lorsque l'on observe que Facebook a racheté progressivement WhatsApp et sa concurrente Instagram, on imagine la quantité phénoménale de données que cette entreprise est capable de posséder et de traiter.

Comment pouvons-nous adapter nos outils de régulation à ce type de mesures et d'évaluation de richesses ? Nous mesurions jusque-là les effets de monopole sur des données économiques. Aujourd'hui, la politique de concurrence doit prendre en compte la détention de données personnelles,

constituent donc un premier axe stratégique en faveur de la compétitivité des activités françaises dans ce secteur. Toutefois, il convient aussi d'engager les entreprises dans une nouvelle logique d'ouverture et de partage de données. Le Gouvernement soutiendra et encouragera

des données par un seul acteur. Ces politiques d'ouverture et de valorisation des données, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont inconcevables sans un cadre protecteur des données personnelles. C'est précisément tout l'intérêt du règlement général de la protection des données, qui entre en vigueur le 25 de ce mois. Il offre aux Européens un niveau de protection inégalée dans le monde, et c'est un atout fondamental pour la France et l'Europe dans la compétition internationale. Les produits et services numériques commercialisés par les Européens sont les seuls à offrir de tels standards de protection sur la vie privée et les données personnelles : il s'agit d'un atout commercial que toutes les entreprises françaises et européennes doivent systématiquement mettre en avant. Les évolutions récentes

« d'outre-mer », membres de l'Union européenne malgré des régimes d'exception de moins en moins protecteurs, deviennent des zones de déversement des trop-pleins de production de la zone Europe. Ces produits arrivent en quantité astronomique et font l'objet d'une grande braderie, aussi bien en qualité qu'en prix. Les producteurs locaux, impuissants, assistent à cette concurrence sauvage de ces productions aidées par les régimes d'éloignement de l'Union européenne, entre autres le Dans ladite « outre-mer », plus encore qu'ailleurs en France, vu la cherté de la vie, la course au moindre coût oriente le choix des consommateurs. Ces déversements sont fréquents, sauvages. Ils n'obéissent à aucune règle, ne sont pas contingentés et surviennent à

a choisi de l'évincer de ses étals au profit d'une banane équatorienne dite « bioéquitable ». Le drapeau bleu-blanc-rouge qui sertissait nos fruits jaunes a été remplacé par le label international Max Havelaar

et environnementales exigeantes. En effet, l'Équateur a obtenu, dans cet accord, de passer d'un tarif douanier de 167 euros par tonne à un tarif de 75 euros par tonne. de 75 euros par tonne. La ministre Annick Girardin et le ministre de l'économie et des finances, qui connaissent très bien ce sujet, plaident auprès du commissaire européen compétent pour que la situation des producteurs de bananes ultramarins soit mieux prise en compte dans le futur accord en 2020. La parole

C'est ce même choix qui prévaut pour l'ouverture à la mondialisation. Le principe d'une économie ouverte n'implique cependant pas une foi inconditionnelle dans le fonctionnement des mécanismes du marché. Il exige au contraire une vigilance constante, pour que le jeu de ces mécanismes puisse être préservé et orienté dans le sens de l'intérêt général. Conçue comme la contrepartie de la libre circulation des marchandises, la politique de concurrence européenne consiste à repérer et à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles concentrations, ententes, abus de position dominante. Cette politique de concurrence a aujourd'hui atteint ses limites et ne peut plus être appréhendée d'une manière purement juridique. Elle doit également être envisagée d'un point de vue économique, social et sanitaire. En ouvrant ses frontières, l'État français participe à la mondialisation de l'économie. Il doit en assumer les responsabilités. À ce titre, il doit assurer la protection non seulement des consommateurs, mais également des producteurs nationaux, qu'ils soient industriels, transformateurs, éleveurs ou agriculteurs. Dans de nombreux domaines, on constate en effet que les produits français se voient imposer des normes très strictes induisant des coûts de production élevés, pour ensuite subir la concurrence de produits importés qui ne respectent pas ces obligations. Cela concerne, par exemple, les normes sanitaires et phytosanitaires, environnementales, sociales, les conditions de travail et les obligations de description des produits à la vente. L'État négocie des accords internationaux qui permettent l'importation de produits ne respectant pas les normes européennes et françaises imposées à nos producteurs. Ces transactions doivent être empêchées ou, à tout le moins, taxées, afin de limiter la concurrence déloyale qu'elles représentent, et faire l'objet d'une information précise auprès du consommateur.

mais j'ai plutôt l'impression d'un fatalisme certain face à la situation qui a été décrite par beaucoup d'intervenants. Pendant ce temps, notre tissu économique se délite, qu'il s'agisse de l'industrie ou de l'agriculture.

C'est sur ces sujets qu'il faut travailler pour éviter un effondrement de notre économie marchande.

handicap en matière de concurrence économique au sein même de l'Union européenne par rapport aux autres pays socialement comparables. À mon sens, ce handicap a deux causes. La première est le niveau des prélèvements obligatoires

Il faut conclure